Monsieur le président,

Cet amendement vise à embrasser les relations intimes qui peuvent exister entre deux individus et à éviter que la relation d'une autorité territoriale ne puisse travailler avec celle-ci au sein de son cabinet. Il serait paradoxal

Les relations privées sont privées ! Je ne vois pas comment le président de la collectivité pourrait être informé, et encore

de chacune des assemblées parlementaires, dans le respect du principe d'autonomie. N'allons pas ajouter et empiler des dispositions législatives qui feraient intrusion dans l'organisation de notre travail, alors que nous sommes si jaloux

! C'est d'ailleurs pourquoi, madame la garde des sceaux, j'insiste tant sur la nécessité de ne pas rendre banale la procédure accélérée. Il faut du temps pour faire des lois

La réserve parlementaire serait un élément de « corruption », les emplois que nous pouvons mobiliser pour exercer notre activité seraient naturellement « fictifs », et les moyens mis à la disposition des parlementaires pour leur permettre d'agir seraient forcément utilisés à des fins qui ne sont pas celles pour lesquelles ils ont été établis ... Tout cela donne une image de la représentation nationale et de la politique absolument catastrophique, qui encourage

menées par leurs propres banques au motif qu'ils sont susceptibles d'être soumis à la corruption ! Nous assistons à une remise en question de la démocratie parlementaire elle-même. C'est vrai ! Je le dis d'autant plus fortement que je suis favorable à des mesures de transparence sur tous les sujets que l'on vient d'indiquer.

en quoi il serait opportun de distinguer entre les petites communes et les communes plus importantes s'agissant de l'objectif d'interdiction des emplois familiaux.

Je vais retirer cet amendement,

n° 176 rectifié. Cet amendement vise à tirer les conséquences des modifications proposées à l'article 4. En effet, la question des emplois familiaux ne saurait résumer à elle seule celle des emplois dits « fictifs », pour lesquels la justice a ouvert un certain nombre de procédures.

non familiaux, alors même qu'il s'agit de rétablir la confiance dans l'action publique. Pourtant, les dispositions du présent article créeront une rupture d'égalité manifeste, contraire à l'objectif initial proposé, sauf à considérer que tous les emplois familiaux sont des emplois fictifs et relèvent des dispositions du code pénal qui les répriment. Les auteurs de cet amendement rappellent à cet égard que les différentes enquêtes en cours, qu'elles en soient au stade de l'instruction ou de l'enquête préliminaire, et dont certaines sont à l'origine du titre III du présent projet de loi, portent notamment sur des faits de « détournements de fonds publics » en ce qu'elles interrogent la réalité des emplois concernés,

Le scrutin est ouvert.

L'application de l'interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours est particulièrement brutale pour les salariés concernés, même si le texte issu de la commission des lois améliore le dispositif envisagé par le Gouvernement.

même si le texte issu de la commission des lois améliore le dispositif envisagé par le Gouvernement. Il nous semble plus juste d'appliquer cette interdiction aux contrats futurs.

Cet amendement présente plusieurs avantages. D'une part, il ne remet pas en cause, contrairement à d'autres, les dispositions du code du travail et ne crée pas de licenciement. D'autre part, il reste conforme à l'esprit du texte du Gouvernement. Pour les sénateurs dont le mandat se termine en 2017, les licenciements s'effectueraient dans les mêmes termes que pour un collaborateur

assurer l'accompagnement vers un autre emploi, nous avons prévu, et c'est la première fois pour des assistants parlementaires qui perdent leur emploi, la possibilité de bénéficier

entre exercer son préavis et percevoir son indemnité compensatrice de préavis. La règle de droit commun s'appliquera. Du coup, l'amendement est déjà satisfait

imaginons même que le Conseil constitutionnel soit saisi -, le délai de cinq mois nous amènera peut-être au-delà du 31 décembre. Exactement ! Il serait donc incompréhensible que je ne retire pas cet amendement.

Il ajoute à la référence aux dispositions du code du travail relatives à la protection des femmes enceintes en matière de licenciement une référence à celles qui concernent les salariés atteints d'une maladie ou victimes d'un accident non professionnel.

Il nous semble donc un peu superfétatoire de les rappeler. Par ailleurs, ce sujet pourrait faire l'objet d'une discussion entre vous lorsque vous évoquerez les règles statutaires applicables aux collaborateurs. Je sollicite également le retrait de ces amendements. Monsieur Détraigne,

des assemblées délibérantes des collectivités et des intercommunalités. On y ajoute parfois les membres de l'assemblée délibérante quand ils sont titulaires d'une délégation de leur président. En ce qui me concerne, j'ai quelques doutes sur cet amendement, qui ne couvre pas ce dernier cas. C'est pourquoi je demande l'avis du Gouvernement, qui permettra, je l'espère, d'éclairer notre débat et de nous prononcer utilement sur cet amendement.

au cours de laquelle il a été demandé aux représentants envoyés par les Français dans les différentes assemblées parlementaires de rendre compte des votes qu'ils avaient exprimés.

Voilà ! Il me paraît tout à fait sage et judicieux que cet usage existe. Votre groupe, monsieur Collombat, comme tous les groupes, a la faculté de demander à tous les parlementaires de s'exprimer sur tout sujet.

... Toujours est-il que je tiens à défendre ici ce droit à demander un scrutin public, pour que chacun d'entre nous doive et puisse rendre compte des votes qu'il a émis en vertu du mandat dont il est le titulaire.

Nous le savons, il y a eu des tarabistouilles dues à la jurisprudence qui permet à certains présidents de groupe de porter 130 ou 140 cartes.

! Nous y sommes d'ailleurs généralement très attachés, parce que c'est aussi une manière de faire respecter les équilibres démocratiques de notre assemblée et d'éviter précisément des votes surprises ou des votes de circonstance, qui eux ne sont pas démocratiques.

Au nom du Sénat de la République, je vous souhaite la bienvenue et je forme des voeux pour que votre séjour en France contribue à renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays.

Cet amendement vise à instaurer de la transparence dans le statut des collaborateurs des groupes parlementaires. En effet, les collaborateurs des parlementaires sont mentionnés, ainsi que leurs activités annexes, dans les déclarations d'intérêts de leur parlementaire. Il serait logique que les collaborateurs des groupes politiques

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

qui n'ont eu de cesse de nous alerter pour demander que le droit commun en matière de licenciement leur soit appliqué. Cet article 6 , adopté sous l'impulsion de notre président rapporteur, constitue un pas important. Je crois pouvoir dire qu'il va dans le sens des revendications qui nous ont été présentées. Toutefois, nous aurions souhaité que le licenciement de nos collaborateurs soit codifié.

personnel. Certains collaborateurs ne se verront donc pas proposer la possibilité de choisir ou non un contrat de sécurisation professionnelle. Nous considérons, pour notre part, qu'il s'agit d'une rupture d'égalité, ce qui ne nous satisfait pas. Certes, le parlementaire employeur est libre de recruter ses collaborateurs, mais le mode de licenciement ne devrait pas être pour lui à la carte.

attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, plan d'épargne entreprise, mutuelle collective, numéro de SIREN -témoignent, nous sommes des « établissements secondaires De plus, il y a quelques points que nous aurions souhaité éclaircir. Les dispositions de cet article 6 sont renvoyées au décret.

toutes les conditions d'exigibilité sont, elles aussi, renvoyées au décret. Nous souhaitons donc que ces points d'incertitude soient levés

ce constat, c'est que les collaboratrices et les collaborateurs parlementaires peuvent, à tout moment, perdre leur emploi en raison d'un décès, d'une non-réélection ou d'une démission du parlementaire employeur.

pouvoir bénéficier, dans cette hypothèse, d'un licenciement pour motif économique. Cependant, force est de constater que cette proposition a été balayée par divers moyens, notamment au nom de l'article 40 de la Constitution. Nous l'avons évoqué hier soir très tard. J'avoue ne pas parvenir à complètement comprendre en quoi ce type de licenciement serait plus coûteux pour nos finances publiques que le licenciement proposé par M. le rapporteur ou que le dispositif actuel. Nos collaboratrices et collaborateurs nous appuient tous et nous aident au quotidien. Si je regrette personnellement, avec d'autres, que le licenciement pour motif économique ait été déclaré irrecevable et soit interdit dans l'usage par l'AGAS, il me semble qu'une solution digne doit être trouvée pour encadrer au mieux la fin de contrat. En ce sens, la possibilité d'un contrat de sécurisation professionnelle doit leur être ouverte. En effet, ce dispositif leur permettra de valoriser les compétences qu'ils ont acquises durant le mandat et de suivre une formation professionnelle pour retrouver rapidement un emploi ou changer de secteur d'activité.

En ce qu'il qualifie la rupture du contrat de travail des collaborateurs parlementaires en cas de fin de mandat de licenciement pour motif économique, entraînant l'application de règles d'indemnisation du chômage plus favorables que celles qui prévalent en cas de licenciement pour motif personnel, cet amendement crée une charge au sens de l'article 40 de la Constitution. » Or cet article 6 , proposé par le rapporteur et voté en commission, concerne les collaborateurs parlementaires qui font l'objet d'un licenciement « pour un motif autre que personnel ». Il se trouve que, pour le moment, le code du travail reconnaît deux types de licenciement, celui pour motif personnel et celui pour motif économique. Je crois que, là, nous nous jouons de mots et je tenais à le dire

pendant douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle ce même collaborateur aurait pu prétendre au titre de l'allocation chômage mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail, à savoir la partie du code du travail qui traite de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. Cette allocation d'assurance chômage prend aujourd'hui le nom d'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Son montant ne peut pas être inférieur à 57 %, ni supérieur à 75 % du salaire journalier de référence : le taux de 57 % correspond à un licenciement pour motif personnel et économique ;

dans nos différents amendements, de codifier le dispositif créé à l'article 6, qui a tous les attraits d'un licenciement pour motif économique, nous agissions dans un souci d'intelligibilité de la loi. Je regrette donc qu'ils aient été jugés irrecevables.

pour procéder au licenciement tel que nous le faisions jusqu'alors, mais assorti des avantages liés au licenciement économique, sans en reprendre toutes les contraintes.

ou en application de l'interdiction des collaborateurs familiaux, un dispositif d'accompagnement renforcé et d'indemnisation améliorée au titre de l'assurance chômage inspiré du contrat de sécurisation professionnelle

pour que le parallélisme des formes soit total avec le CSP, il convient de préciser le dispositif prévu par la commission des lois sur deux points. Il s'agit, d'abord, de préciser la façon dont le dispositif est proposé au collaborateur licencié. Le présent amendement prévoit, comme pour le CSP, que ce soit le parlementaire employeur qui le propose à son collaborateur. Il s'agit, ensuite, de préciser les conséquences de l'acceptation par le collaborateur du dispositif. Comme dans le cadre du CSP, le présent amendement prévoit que l'acceptation du dispositif emporte la rupture immédiate du contrat de travail et le versement par l'employeur de l'équivalent de l'indemnité de préavis à Pôle emploi pour le financement de l'accompagnement du salarié et de la majoration de son indemnisation.

monsieur le rapporteur, de la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis. D'autre part, Pôle emploi fait apport des financements nécessaires pour assurer la sécurisation de son parcours professionnel. Pendant cette période, la question de l'indemnisation qui se met en place est tout naturellement réglée par Pôle emploi.

au collaborateur. Rien ne sera imposé. Le collaborateur choisira telle ou telle indemnisation. Bien sûr, après, comme pour tout, c'est l'AGAS qui apporte la

-préparer le « concours de l'ENA ». Cela m'a un peu étonnée, et je suis donc allée consulter le site de l'AGAS. J'ai bien vu qu'il existait un cycle de perfectionnement organisé par l'ENA, mais à destination des collaborateurs

cette disposition devient sans objet. Je crois qu'il faut choisir : ou bien on fait un troisième concours- ce qui est très bien -, ou bien on ouvre le concours interne, ce que M. Zocchetto et Mme Assassi nous ont proposé et que nous avons admis hier, mais on ne peut tout de même pas retenir les deux ! Peut-être ce débat va-t-il cependant se poursuivre. Je sais d'ailleurs que les représentants des fonctionnaires de cette maison

pour des raisons que certains comprendront ici. C'est pourquoi je vais, bien sûr, retirer cet amendement, mais en souscrivant aux propos de notre président-rapporteur,

de la procédure accélérée ne lui impose nullement de ne prévoir qu'une lecture par assemblée. Je ne vois pas pourquoi nous préjugerions de sa décision, qui peut fort bien consister à permettre au débat de se poursuivre dans l'intérêt de la loi.

ils incitent des petits partis, parfois des pseudo-partis, à présenter un maximum de candidats. Par cet amendement, nous proposons que ces aides soient attribuées à un parti lorsque cinquante de ses candidats, comme c'est déjà le cas, ont obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés,

une aide publique au financement. En effet, ces seuils sont trop bas : ils peuvent permettre à certains partis ou groupements politiques, voire à des partis globalement fictifs, de capter des subventions publiques sans remplir effectivement les fonctions à travers cette mesure, notre objectif est de subordonner le financement public à trois conditions : avoir un réel objet politique, rassembler des militants et soutenir des candidats aux élections locales et nationales. L'amendement

Si nous plaçons la barre trop haut, nous écartons de tout financement public des courants de pensée qui ont une audience réelle dans l'opinion, même si ce sont des partis minoritaires.

permet de poser une condition d'audience pour l'accès au financement public, mais exige qu'on respecte le pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie. Tout cela me paraît être de pur bon sens. Nous avons débattu en commission pour déterminer à partir de quel seuil

Par conséquent, la demande qui nous est faite à travers ces amendements est tout à fait légitime. Néanmoins, je ne voudrais pas que le Sénat se prononçât à l'aveugle,

auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, pour lui demander si nous pouvons trouver un terrain d'entente à partir de ces projections afin de déterminer exactement où placer le seuil.

de supprimer l'aide publique à Debout la France, à l'Alliance écologiste indépendante ou même au Parti radical de gauche.

Monsieur le président, peut-être nos collègues voudront-ils abaisser les seuils qu'ils ont déterminés dans leurs amendements, auquel cas la commission pourrait reconsidérer l'avis que j'ai donné, qui reposait sur celui du Gouvernement. La

de vote. Personne ici ne souhaite la disparition du financement public des partis

du financement des partis politiques. Pour financer leurs dépenses, les partis politiques reçoivent une aide de l'État. Pour certains d'entre eux, cette aide constitue la principale source de financement. En contrepartie, les dons des personnes morales sont frappés d'interdiction. Les crédits destinés à être versés aux partis et groupements politiques sont inscrits, chaque année, en loi de finances. Ils sont répartis entre les partis politiques pour pour moitié à raison de leurs résultats au premier tour des élections législatives. Cette première part bénéficie aux partis ayant présenté, dans au moins cinquante circonscriptions ou dans au moins un département ou une collectivité d'outre-mer, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés. Elle est réduite en cas de méconnaissance des règles favorisant la parité entre les femmes et les hommes. L'autre moitié est répartie aux partis représentés au Parlement, en proportion du nombre de députés et sénateurs. Seuls les partis bénéficiant de la première fraction sont éligibles à la seconde. Si les règles instituées par la loi du 11 mars 1988 constituent une avancée, le mode de répartition n'est pas satisfaisant. Il contribue à renforcer le bipartisme et reproduit à l'échelle du financement des organisations politiques les distorsions introduites par les modes actuels de scrutin. Au cours de la dernière législature, les deux principales formations politiques ont ainsi touché près de 70 % de l'ensemble de l'aide publique, alors qu'elles avaient obtenu aux élections législatives de 2012 57 % des suffrages exprimés au premier tour. En l'absence de scrutin proportionnel, le fait d'attribuer la moitié de l'aide en fonction du nombre de députés et de sénateurs représente donc une anomalie. Afin de renforcer l'équité du dispositif, les auteurs de cet amendement proposent, conformément à la proposition de loi déposée par nos collègues à l'Assemblée nationale, d'établir de nouvelles règles de répartition de l'aide publique donnant plus de poids à la fraction assise sur les suffrages exprimés en faveur de chaque parti. Nous préconisons que le montant de l'aide publique soit désormais divisé en deux fractions inégales : l'une, correspondant aux trois quarts du montant total, destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats au premier tour des élections législatives

les effets du scrutin majoritaire sur le financement des partis politiques, alors que l'enjeu est précisément de permettre à des partis faiblement représentés, voire pas représentés du tout, de participer quand même au débat démocratique grâce à des financements publics.

Leconte. La loi du 11 mars 1988 exige que chaque parti politique recueille les dons dont il est bénéficiaire par l'intermédiaire d'un mandataire, qui peut être une personne physique ou une association de financement.

La commission n'a pas de conviction fermement arrêtée dans ce domaine : elle s'en est tenue au projet de loi du Gouvernement. J'ai bien entendu l'exposé des intentions de l'auteur de cet amendement. Je me souviens aussi de ce que le président de la Commission

défendre M. Jean-Pierre Sueur. L'objectif est d'éviter toute ambiguïté en interdisant complètement les prêts consentis par des personnes physiques à des partis politiques. On peut toujours trouver des moyens pour mieux les contrôler, mais on sait bien que la seule solution pour en finir avec ce système de prêts qui se transforment en dons est d'interdire complètement les prêts. Par conséquent, je me rallie à l'amendement n° 117 et je retire le

Si l'on ne peut interdire les prêts entre ces différentes entités juridiques, on peut interdire à ces formes de mini-banques privées de la vie politique de faire des bénéfices en se rémunérant sur les prêts qu'elles accordent.

concernant le financement des campagnes électorales, à l'article 9 du présent projet de loi. Quel est

une obligation de publicité par cette instance des donateurs de plus de 2 500 euros. L'exigence de transparence conduit ainsi à rendre accessibles à tous, et non pas seulement à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ces informations importantes pour la compréhension des liens d'intérêts et de finances entre un candidat ou un parti politique et des personnalités influentes. Peut-être se souvient-on ici

dans lesquelles il faisait référence à la levée de fonds du président Macron à la City, à New York, parmi des banquiers et autres puissants de ce monde et s'interrogeait sur cette problématique. Nous partageons sa volonté de limiter la porosité entre la finance et la politique, même si la politique a besoin de financements. C'est

et ce depuis maintenant 128 ans. Cette règle a été inventée pour permettre à nos concitoyens d'échapper à toute pression.

à la divulgation d'une information qui relève strictement de sa vie privée et des choix qu'il accomplit en conscience

est ainsi libellé : La parole est à M. Jean-Pierre Grand. Avec les établissements de crédit et sociétés de financement, les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique et des candidats aux élections. Afin d'éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d'interdire la fourniture de prestations surfacturées d'un parti ou groupement politique à un candidat lors d'une campagne électorale et des partis et groupements politiques entre eux. Quel est l'avis de

79 est retiré.

à savoir la perte de la possibilité de financer la campagne électorale d'un candidat ou d'un autre parti politique, n'est toujours pas inscrite dans la loi. Comme le soulignait la

est à M. Jean-Pierre Grand. L'article 9 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats a permis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de moduler les sanctions et leur durée en cas de manquement aux obligations comptables pour une meilleure proportionnalité entre les motifs du constat et ses conséquences juridiques. Cette disposition est conservée dans la nouvelle rédaction de l'article 11-7 proposée à l'article 8 actuelles dispositions relatives à la sanction du non-respect des obligations comptables semblent ne pas atteindre complètement l'objectif. En effet, certaines formations politiques défaillantes peuvent, peu après la décision les concernant, créer un parti politique « frère dont la dénomination est très proche et qui est uniquement destiné à se substituer l'année suivante à la formation en cause pour l'encaissement des dons et cotisations. Les fonds ainsi perçus ouvrant droit à la réduction d'impôt au bénéfice des sympathisants et adhérents, la formation nouvellement créée peut ensuite en toute légalité les reverser au profit du parti pour lequel un manquement avait été constaté. Ce constat illustre la difficulté pour le législateur de définir une sanction adéquate et efficace à l'encontre des partis politiques qui ne respecteraient pas les obligations prévues par la loi sur la transparence financière. Sans Sans remettre en cause la liberté constitutionnelle de création et d'organisation des partis politiques, il est proposé d'interdire à un parti ou groupement politique sanctionné de recevoir des contributions financières d'autres partis ou groupement politiques. Il s'agit là de répondre à une de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, notamment dans son seizième rapport d'activité,

monsieur le président.

des dispositions des articles 8 à 10 de la loi de 1988 et du bénéfice de la réduction d'impôt prévu à l'article 200 du code général des impôts. La durée de ces sanctions initialement fixées à un an a été portée à trois ans par la loi du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats. Compte tenu de tous ces éléments, il ne paraît pas opportun de changer la loi. La parole

L'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 prévoit que les partis et groupements politiques ont l'obligation de tenir une comptabilité et de déposer des comptes certifiés, lesquels sont contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La loi du 11 mars 1988 ne donne aucune définition des partis et groupements politiques. Son champ d'application résulte de l'économie générale du dispositif de transparence du financement de la vie publique politique telle qu'elle a été interprétée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. En l'état du droit, les les obligations comptables s'imposent, d'une part, aux partis et groupements politiques qui bénéficient d'un financement public, d'autre part, à ceux qui se soumettent au dispositif prévu par les articles 11 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988. Ce dispositif repose sur le recours à un mandataire et sur la mise en oeuvre d'un cadre strict de financement. En contrepartie, les partis et groupements politiques peuvent notamment recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt et contribuer au financement des campagnes électorales ou d'autres partis. Les obligations comptables prévues par la loi du 11 mars 1988 et le contrôle de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques n'ont de sens que pour ces seuls partis et groupements politiques. Étendre les obligations comptables à l'ensemble des partis et groupements politiques serait de nature à remettre en cause l'équilibre du dispositif de transparence du financement de la vie politique issu de la loi de 1988 et validé par le Conseil constitutionnel au regard de l'article 4 de la Constitution. Compte tenu des sanctions administratives et pénales dont est assorti le non-respect des obligations comptables prévues par l'article 11-7, il est indispensable d'éviter toute ambiguïté ou difficulté sur leur champ d'application.

et n'étant pas propriétaires de leur local. Ainsi, l'amendement prévoit qu'un décret fixera les conditions détaillées d'application de cette disposition, qui ne concernera que les organisations territoriales du parti ou groupement politique ayant des revenus ou des actifs significatifs. Quel

Cet amendement vise à exclure de la présentation des comptes consolidés des partis les comptes des petites structures territoriales. L'inclusion dans la comptabilité des partis et groupements politiques des comptes de toutes les organisations territoriales du parti politique est un facteur fondamental d'amélioration de la transparence et de la traçabilité de leurs ressources.

à M. Jean-Pierre Grand. Actuellement, les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et les partis ou groupements politiques peuvent les conserver d'un mandat à l'autre. Certains partis ou groupements ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant de très nombreuses années, ce qui peut engendrer des situations susceptibles de remettre en cause l'impartialité ou l'indépendance des commissaires aux comptes désignés. Cet à introduire une obligation de rotation des commissaires aux comptes sur le modèle des dispositions prévues dans le code de commerce pour les commissaires aux comptes des associations faisant appel public à la générosité. aux comptes ne pourraient certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs et seraient remplacés tous les six ans. Il s'agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Quel est

des informations importantes, notamment le nom des principaux dirigeants, nécessaire pour identifier le parti, les flux financiers avec d'autres partis- information nécessaire pour déceler d'éventuels circuits financiers ou détournement de la loi, par exemple par des partis qui ne se regrouperaient que pour bénéficier de financements publics -, ou encore le nombre d'adhérents et de cotisants pour juger du poids réel du parti. Il est également proposé que la transmission et la publication de ces données se fassent au format ouvert pour être plus facilement utilisées, comme l'a déjà proposé la commission des lois. Le mode de publication de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'est plus adapté aux réalités actuelles. Dès lors, la transmission des annexes se ferait également en.

de s'assurer de la transparence financière et de la régularité des comptes, non de contrôler l'activité d'un parti politique. Nous ne pouvons prendre le risque constitutionnel

selon les règles de droit commun. Je ne comprends pas que le Gouvernement puisse vouloir restreindre le champ de l'information des Français

sur l'amendement n° 202 rectifié. En effet, la loi du 11 mars 1988 prévoit déjà la publication d'un certain nombre de documents et d'informations relatifs aux comptes des partis et à leurs sources de financement. Des remontées d'informations très précises sont prévues, notamment pour les dons, les cotisations et les emprunts. Cette disposition permet de garantir de manière suffisante la transparence vis-à-vis des citoyens, ainsi que l'effectivité du contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. De plus, la commission des lois a adopté un amendement tendant à prévoir la mise à disposition des comptes des partis en. La

quatre sénateurs et deux députés n'ont pas indiqué de rattachement. Lorsqu'un parlementaire n'indique pas de rattachement, aucune disposition ne traite le problème des sommes auxquelles un parti politique aurait eu droit s'il en avait choisi un. C'est précisément, si je l'ai bien compris, tout l'intérêt de votre amendement que de traiter cette question

depuis la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, proscrit tout lien financier entre personnes morales et partis politiques. Par analogie, le présent projet de loi interdit également les prêts des personnes physiques à destination d'une campagne électorale. Il prévoit cependant des exceptions à cette interdiction. Ainsi, les établissements de crédit et les partis politiques pourraient consentir des prêts à un candidat. Notre amendement a pour objet d'étendre l'interdiction faite aux personnes morales de financer les campagnes électorales aux partis politiques eux-mêmes.

Nous souhaitons ainsi inciter les partis, qui ne pourraient désormais plus consentir de prêts aux candidats, à créer une structure indépendante qui pourrait, elle, contrairement aux partis en vertu de l'article 4 de la Constitution, être contrôlée. Cet amendement est donc non pas un non ferme et définitif aux prêts des

M. Jean-Pierre Grand. La jurisprudence du Conseil d'État a établi un lien entre le respect des obligations comptables et le financement des campagnes électorales en privant le parti défaillant de cette possibilité. En effet, en perdant le bénéfice de certaines dispositions de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un parti ou groupement politique redevient une personne morale non autorisée à participer au financement d'une campagne électorale. Il est donc proposé de codifier cette interdiction de financement, qui sera sanctionnée

Si l'encadrement de l'activité de prêt peut être discuté, l'interdiction pour un parti politique de soutenir financièrement un candidat se heurterait, mes chers collègues, à l'article 4 de la Constitution, qui prévoit

adopté, cet amendement risquerait de heurter les engagements internationaux et européens de la France, notamment ceux qui assurent une liberté de prestation de services au sein de l'Union européenne. Pour cette raison, la commission y est défavorable. L'amendement n° 81 de M. Grand

La confiance dans l'action publique repose également sur la bonne utilisation de l'argent public, notamment dans le cadre des élections. Il convient de rappeler que l'État participe au financement des campagnes électorales à la fois par le remboursement d'une partie des dépenses de campagne- c'est l'apport personnel du candidat -et par la délivrance d'un avantage fiscal aux donateurs, à hauteur de 66 % du montant du don déductible des impôts, ce qui n'est pas rien. L'article 112 de la loi 2011 de finances pour 2012 a réduit de 5 % les taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne. Il est ainsi passé de 50 % à 47,5 %.

Chaque fois que l'on abaisse la part des dépenses susceptibles d'être prises en charge par l'État, on rend en réalité le candidat plus dépendant du financement de son parti, si lui-même n'a pas de fortune personnelle,

des candidats qui relèvent d'un grand parti politique venant de gagner des élections nationales et dont les caisses sont renflouées du fait de cette victoire, et de rendre plus vulnérables

madame la ministre, Pour autant, l'objet de ce texte n'est pas de diminuer les dépenses de campagne, et il n'est pas non plus d'assécher les sources de financement des candidats aux élections. L'objet est de mieux encadrer le financement des campagnes électorales et d'en assurer la transparence.

et des partis et groupements politiques. La perspective d'un remboursement d'une partie des dépenses électorales est de nature à favoriser l'octroi d'un crédit. Par ailleurs, le plafond des dépenses de campagne n'est plus réactualisé à la hausse depuis un décret de 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales pour tenir compte de l'inflation. Ajouter à ce gel une diminution du plafond des dépenses et des remboursements porterait selon nous une atteinte démesurée au financement de la vie démocratique dans notre pays. Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

des services de l'État dans l'acheminement de la propagande électorale officielle.

à des élections nationales. Ainsi, si vous avez été candidat aux élections législatives en 2012, vous entrez une bonne fois pour toutes, pour les établissements bancaires, dans la catégorie des personnes politiquement exposées. Nous avons pensé, à la commission des lois, que le risque était grand de voir les organismes bancaires mettre en cause l'existence même du compte d'une personnalité politiquement

nous appuyer sur l'existence du compte personnel du candidat pour imposer à la banque de lui ouvrir un compte en tant que candidat. À cette solution, nous avons préféré une formule qui nous paraît opérationnelle

est que la banque s'abstient de toute réponse à réception de la demande d'ouverture du compte. Dès lors, les dispositions qui permettent déjà de contraindre la banque à ouvrir le compte de campagne ne trouvent pas à s'appliquer, car la Banque de France ne peut pas être saisie.

l'adoption de cet amendement risque d'être contre-productive et de rendre difficile l'ouverture d'un compte personnel pour les mandataires. Nous jugeons préférable de nous en tenir aux modalités de droit au compte prévues par le code électoral,

Je rejoins les propos de M. le rapporteur, qui, à plusieurs reprises dans ce débat, a insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions d'accès des mandataires des candidats et partis à un compte bancaire et aux prestations bancaires de base. Le Gouvernement propose donc deux modifications au texte adopté par la commission. D'une part, pour les prestations de base que l'établissement de crédit est tenu de proposer, le renvoi à un décret ne paraît pas utile dès lors que le code monétaire et financier définit déjà ce que sont ces prestations de base. Le renvoi au droit commun est suffisant. Les partis et candidats auront notamment droit, sans limitation et gratuitement, aux prestations de dépôt d'espèces et d'encaissement de chèques, prestations particulièrement importantes, en particulier pour les dons. D'autre part, et cela apparaît tout à fait essentiel, il est nécessaire d'harmoniser les conditions de clôture des comptes à l'initiative de l'établissement,

Cet amendement a pour objet d'introduire un peu de souplesse dans les règles de financement des des campagnes électorales. Afin que les comptes de campagne soient tenus de façon rigoureuse, légitime et juste, le législateur exige depuis quelques années une stricte séparation entre séparation entre l'ordonnateur- le candidat -et le payeur- le mandataire de la campagne. Or, à l'usage, il apparaît qu'un assouplissement, d'ailleurs limité, serait utile.

et que l'on peut soupçonner que la non-déclaration dans le compte de campagne des menues dépenses a pour objet de ne pas dépasser le plafond, elle sera plus sévère.

Cet amendement vise à faciliter le travail de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en lui permettant de recourir aux services de

C'est une bonne chose. Chacun sait que l'accès au financement et notamment au crédit peut être une démarche semée d'embûches pour les partis politiques et pour les candidats aux élections. Il s'agit là d'une entrave au bon déroulement de la vie démocratique de notre pays et d'un facteur d'inégalités entre les candidats. le rapporteur, la commission a modifié la dénomination de « médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques » en « médiateur du financement des candidats et des partis politiques ». Nous approuvons l'élargissement des missions de ce médiateur. Notre seule interrogation

une véritable question qui ne peut être laissée à la seule appréciation du secteur bancaire privé de notre pays. Pour cette raison, nous regrettons la suppression, à l'article 12, de la banque de la démocratie. Certes, le Conseil d'État a émis des réserves quant au fonctionnement de cette instance, et de nombreuses incertitudes planaient sur ce dispositif. Pour autant, il est aujourd'hui nécessaire de réguler l'accès au financement des organisations politiques comme des associations. Nous ne souscrivons pas à l'argument selon lequel « seule une insuffisance avérée du marché de l'accès au crédit pour les candidats et les partis politiques, après intervention éventuelle du médiateur, pourrait justifier sous quelque forme que ce soit une intervention sous la forme d'une structure dédiée ». Au contraire, nous pensons qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir l'accès de tous au financement. C'est une question éminemment démocratique. Nous regrettons donc largement cette suppression, même si, je le répète, cette création passait par l'habilitation du Parlement au Gouvernement à agir par voie d'ordonnance. Nous espérons évidemment que cette discussion reprendra.

en particulier l'extension des missions du médiateur aux litiges relatifs à l'ouverture d'un compte bancaire et à l'accès aux prestations bancaires de base. Pour autant, je ne peux soutenir ni le changement de nom du médiateur ni l'insertion du dispositif dans la loi du 11 mars 1988. il nous semble que la mission centrale du médiateur demeure l'accès au crédit. En conséquence, il nous paraît indispensable que les parties prenantes puissent identifier aisément leur interlocuteur privilégié dans ce domaine : voilà pourquoi le nom de « médiateur du crédit » nous semble plus clair. De plus, le nom de « médiateur du financement » et l'insertion du dispositif dans la loi de 1988 seraient, à nos yeux, sources d'ambiguïtés : le médiateur n'a pas vocation à intervenir sur les autres modes de financement des partis et des candidats, modes de financement que l'on sait très variés. Enfin, le mode de nomination du médiateur doit être clair. La procédure prévue par l'article 13, alinéa 5, de la Constitution offre offre toutes les garanties nécessaires pour assurer la désignation d'un médiateur qualifié et indépendant. Le gouverneur de la Banque de France émettra un avis simple, alors que, comme vous le savez, les assemblées parlementaires pourront s'opposer à la désignation du médiateur. L'établissement d'une liste limitative de candidats par le gouverneur de la Banque de que prévoit le texte adopté par la commission des lois, ne paraît pas compatible avec cette procédure. C'est pourquoi, de notre point de vue, il conviendrait de revenir sur ce point à la rédaction initiale du présent projet de loi.

Sur cet article, nous défendons la position de la commission, mais nous souhaiterions également revoir le dispositif de nomination du médiateur du financement. du médiateur du financement. Dans le projet de loi initial, le médiateur était nommé pour un mandat de six ans, par décret du Président de la République, après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, conformément à la loi organique du 23 juillet 2010, et après avis du gouverneur de la Banque de France. La commission a revu ce mode de nomination pour donner un réel pouvoir propositionnel au gouverneur de la Banque de France. C'est effectivement un pas positif, à ceci près que le gouverneur de la Banque de France est lui-même nommé par le Président de la République Pour notre part, nous contestons le fait que cette nomination soit liée à un décret du Président de la République. Nous estimons que ce dispositif contribue à l'hyperprésidentialisation du régime, que nous contestons

nous nous sommes un peu inspirés des modalités de nomination des magistrats du siège. Nous avons estimé que, si le gouverneur de la Banque de France fait une proposition, la procédure lie davantage le Président de la République. Mais il ne faut pas trop le lier non plus. Nous avons donc prévu que le gouverneur de la Banque de France fasse la proposition de trois noms. Parmi ces derniers, le Président de la République choisira de désigner un médiateur pressenti, lequel se présentera devant les commissions des lois

électorales, le recours à l'emprunt bancaire est en recul. Il représentait 35 % du financement des candidats à l'élection présidentielle et 25 % du financement des candidats aux élections législatives en 2012.

Une structure de financement des candidats apparaît donc comme une réponse indispensable pour pallier les carences du financement bancaire privé.

parce qu'elle prévoit plusieurs options. Elle comporte cependant les dispositions nécessaires pour assurer le respect de l'article 38 de la Constitution, comme l'a d'ailleurs précisé le Conseil d'État dans son avis. L'habilitation prévoit que la structure de financement interviendra en cas de défaillance avérée du marché et, le cas échéant, après intervention du médiateur. La banque de la démocratie pourra accorder des prêts, des avances ou des garanties. l'amendement présenté par le Gouvernement tend à resserrer le champ de l'habilitation au financement des campagnes électorales présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes. La banque de la démocratie pourra être un établissement doté de la personnalité morale, adossé à un établissement de crédit existant, ou bien prendre la forme d'un mécanisme de financement spécifique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire devant vous une mission va être confiée en ce sens à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration. Ainsi pourra-t-on déterminer la forme la plus adéquate de cette structure pour qu'elle puisse atteindre au mieux les buts qui lui sont fixés. Par la même occasion, les conditions de sa mise en place l'habilitation précise que les règles de fonctionnement de la structure devront garantir l'impartialité des décisions qui seront prises, de manière à préserver le pluralisme de la vie politique et la viabilité financière du dispositif mis en place. Comme le précise l'étude d'impact, les décisions pourront être prises par une autorité collégiale ne recevant aucune instruction du Gouvernement non plus que d'une autre autorité, afin de préserver l'indépendance de la banque de la démocratie. Les décisions de la banque pourront se fonder sur les perspectives raisonnables de remboursement, reposant elles-mêmes sur des critères objectifs tels que, par exemple, le patrimoine du demandeur ou l'existence de garanties et de sûretés. Concrètement, le critère d'appréciation appliqué par la banque de la démocratie devra être la solvabilité. Ce critère permettra également d'objectiver le cadre d'intervention de la banque. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, cette demande d'habilitation n'est pas la conséquence d'une quelconque impréparation du Gouvernement,

Le Gouvernement souhaite disposer des moyens d'instituer une banque de la démocratie. Cette instance nous semble totalement indissociable des autres mesures réformant le financement de la vie politique, que vous examinez aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous propose de rétablir l'article 12 du présent projet de loi.

le résultat de l'étude qu'il a confiée conjointement à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration. Nous vous faisons réellement crédit des intentions qui sont les vôtres pour améliorer le financement des campagnes électorales et nous sommes tout à fait prêts à débattre avec vous. Cependant, dans ce domaine hautement dérogatoire aux droits du Parlement,

bien, vous n'avez pas matériellement eu le temps d'aller plus loin. Vous avez sans doute besoin d'être davantage éclairée avant de pouvoir nous éclairer vous-même, mais, dès lors que nous ne sommes pas suffisamment éclairés, nous ne pouvons vous déléguer le pouvoir

dédiée au financement de la vie politique soit indispensable, j'en suis absolument persuadé.

ont du mal à obtenir les prêts nécessaires pour financer leur campagne électorale. Nous en faisons encore l'expérience à quelques semaines des élections sénatoriales : nous savons d'ores et déjà

Monsieur le président, en application de l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, je demande l'examen en priorité de l'amendement n° 294 de la commission et du sous-amendement n° 295 dont il fait l'objet.

de l'utilisation de l'argent public par d'autres acteurs de la société. On ne parle ainsi jamais de moraliser la vie économique.

il s'agit des frais liés à la permanence et à l'hébergement du sénateur, des frais de déplacement du sénateur et de ses collaborateurs, des frais de documentation et de communication, des frais de représentation et de réception, des frais de formation du sénateur et de ses collaborateurs et de la participation aux dépenses de fonctionnement d'un groupe parlementaire. Aucune dépense n'entrant pas dans une

sur la prise en charge des frais de mandat de la manière la plus sereine, compte tenu de la réglementation très précise qui existe dans notre assemblée. Je sais d'ailleurs que, dans ses travaux préparatoires, le Gouvernement s'est largement inspiré- il pourra le confirmer -des règles posées par le Sénat

Vous avez également demandé que les frais de mandat soient remboursés

de ce remboursement et l'ensemble des modalités de fonctionnement de la prise en charge des frais de mandat devaient être déterminées par le bureau de chacune des deux assemblées. Toute autre position serait d'ailleurs inconstitutionnelle : il y a une limite à l'intrusion possible du législateur dans le fonctionnement de nos assemblées.

avons considéré que faire du remboursement la modalité unique de prise en charge des frais de mandat était beaucoup trop restrictif et risquait d'entraîner des contraintes bien trop fortes pour l'exercice de notre fonction.

nationale, laquelle dès lors ne se sentira nullement liée par le vote que nous aurons émis. Je souhaite, mes chers collègues, que le Gouvernement défende la position qui aura été débattue au Sénat sur ces points essentiels, car sinon nous risquons

: si l'Assemblée nationale est en désaccord avec le Sénat, le Gouvernement sera conduit à lui donner le dernier mot, et tout le travail patient que nous avons accompli n'aura servi à rien. Ces raisons politiques me paraissent suffire à justifier que j'aie recherché un accord avec le Gouvernement.

l'indemnité représentative de frais de mandat, dont j'ai rappelé à quel point elle était déjà encadrée. Telle n'était pas la volonté de la commission des lois. En revanche, nous avons insisté très fermement sur la nécessité de prévoir trois modalités de prise en charge des la prise en charge directe et le remboursement. Ce point me paraît absolument essentiel. Le Gouvernement, à la suite de nos discussions, a accepté que le texte

du fait d'une probable déperdition (absence de demande de remboursement ou perte de justificatif) ». Je ne sais si c'est cette finalité qui est recherchée, mes chers collègues, mais sachez en tout cas que cela figure dans l'étude d'impact

Mes chers collègues, je vous demande donc, en connaissance de cause, d'adopter ce sous-amendement pour limiter les effets induits que j'ai essayé de décrire rapidement.

de nos collaborateurs, etc. Cet amendement tend donc à remplacer le système proposé de remboursement des frais, qui imposerait aux parlementaires de faire des avances importantes et exigerait la mise en place d'une nouvelle organisation administrative lourde et coûteuse, par un mécanisme d'avances mensuelles, assorti de l'obligation de tenir une comptabilité faisant l'objet de contrôles aléatoires, à l'instar des contrôles fiscaux pour les citoyens. La transparence souhaitée serait ainsi obtenue par des moyens mieux adaptés.

dont on n'ose pas souvent parler, est de maintenir un minimum d'attractivité et d'indépendance à la fonction parlementaire,

donc été décidé de supprimer l'IRFM, pour toutes les raisons qui ont pu être explicitées. Le dispositif figurant dans le projet de loi initial reposait sur les trois principes

Il s'agit là de respecter la séparation des pouvoirs et l'autonomie des assemblées, ce qui conduit également, selon nous, à écarter l'intervention d'un organisme extérieur comme au Royaume-Uni. Vous avez proposé, monsieur le président Bas, qu'il revienne aux bureaux des assemblées de définir ces conditions, après avoir consulté l'organe de déontologie. Naturellement, le Gouvernement n'est absolument pas en désaccord avec cet aspect de l'évolution du texte

entre l'adoption par la commission des lois de la nouvelle rédaction de l'article 7 et hier soir, des échanges extrêmement riches. À cet égard, je tiens à remercier très sincèrement le président de la commission des lois pour la

Ainsi, l'IRFM sera supprimée à compter du 1 janvier 2018, pour être remplacée par un système de remboursement sur justificatifs.

hors IRFM. Par ailleurs, une solution sera apportée pour que les parlementaires n'aient pas à avancer certaines dépenses dans un certain nombre de cas. Je ne méconnais pas les modifications que cette mesure entraînera pour la Haute Assemblée, mais je suis certaine qu'elles sont surmontables. Il appartiendra aux bureaux des assemblées d'organiser concrètement ces dispositifs, en toute transparence et après avis de l'organe de déontologie. Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 294. S'il est adopté, les amendements n 214 et 213, que le Gouvernement avait déposés avant nos échanges fructueux,

monsieur le rapporteur,

des modalités de la prise en charge des frais de mandat. Il aura le choix entre trois formules : le remboursement, la prise en charge directe ou l'avance. Dans les trois cas, des justificatifs

que nous serons en mesure d'évaluer réellement les coûts de gestion pour nos assemblées. Actuellement, comme nul ne sait

il est évident que passer, comme cela pourrait être le cas dans une entreprise, d'un système de forfait à un système de prise en charge sur justificatifs a un coût.

évaluer. Le sous-amendement très ingénieux de notre collègue questeur Jean-Léonce Dupont, qui vise en réalité peu ou prou à rétablir la rédaction initialement proposée par la commission des lois,

Cependant, en n'explicitant pas ce que recouvre la notion de prise en charge, comme nous avons précisément voulu le faire pour rassurer le Gouvernement, il ne nous garantit pas

devant les Français le problème de la rémunération de leurs élus nationaux, de leurs représentants qui expriment la souveraineté du peuple français

que de décider nous-mêmes du montant de nos rémunérations, car il appartient aux Français de dire quelle valeur ils attachent au travail de leurs représentants,

je propose, en accord avec le Gouvernement, un autre système de prise en charge des frais de mandat que l'incorporation de l'indemnité représentative de frais de mandat aux revenus du parlementaire, je ne puis approuver cet amendement, d'autant que,

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

La séance est suspendue.